2017. Si cette évolution législative apparaissait souhaitable pour lutter contre des comportements peu civiques et dangereux qui avaient été constatés, son application pose en revanche de grandes difficultés pratiques, comme le font remarquer certaines associations d'automobilistes.

Ainsi, de nombreux particuliers se voient adresser depuis le 1 janvier 2017 des amendes au montant très important, alors qu'ils ne sont pas concernés par les dispositions adoptées par la représentation nationale. M. Botrel s'interroge sur les raisons d'un tel résultat ; il souhaite que soit respecté l'esprit de la loi votée

Comme vous le savez, l'obligation de désignation s'imposait déjà aux représentants légaux de personnes morales avant le 1 janvier 2017. Le changement que constitue l'envoi d'un avis de contravention pour non-désignation permet de sanctionner un comportement qui, avant cette date, était déjà contraire aux obligations des représentants légaux et aux objectifs de la sécurité routière. Depuis le 1 janvier 2017, les personnes morales dont le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis une infraction au volant d'un véhicule leur appartenant ou qu'elles détiennent reçoivent un avis de contravention pour non-désignation. L'envoi de ce nouvel avis de contravention doit mettre fin à la situation qui voit certains contrevenants ayant commis une infraction au volant d'un véhicule professionnel échapper au retrait de points.

routière. Dès lors qu'un véhicule est enregistré dans le système d'immatriculation des véhicules au nom d'une personne morale, entraînant l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom, son représentant légal a l'obligation de désigner le conducteur qui commet une infraction au volant de ce véhicule. Ni le fait que la personne morale porte le même nom que son représentant légal ni celui que ce représentant est le seul à conduire le véhicule ne sauraient l'exonérer de se désigner en tant que conducteur. Les avis de contravention envoyés aux représentants légaux ne leur sont pas nommément adressés. Y figurent seulement la mention de la qualité de représentant légal du destinataire de l'avis, celle de la raison sociale de la personne morale qu'il représente, ainsi que l'adresse de cette dernière. Afin de faciliter les démarches des représentants légaux, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ou ANTAI, a procédé récemment à l'adaptation des documents qu'elle leur envoie dans le cadre du contrôle automatisé.

l'alimentation. Monsieur le ministre, l'agriculture française présente de nombreux atouts tant économiques que sociétaux. Le Gouvernement et sa majorité ne semblent cependant pas en être vraiment convaincus.

Chacun appréciera ; il était important à mes yeux de le rappeler. L'indépendance et la sécurité alimentaire constituent des enjeux stratégiques aux échelons tant européen que français face à un accroissement de la demande en production agricole et, notamment, végétale, dans un contexte d'augmentation de la population mondiale. Si le climat tempéré de notre pays constitue un atout pour la diversité de nos productions, il est également source d'une forte diversité des bioagresseurs des cultures : ils sont plus de 10 000, évoluent et s'adaptent en permanence. Dans ce contexte évolutif, monsieur le ministre, la santé des plantes est un enjeu au même titre que la santé humaine ou animale. Pour y répondre, limiter les dégâts sur leurs cultures et satisfaire aux exigences des marchés, les agriculteurs ont besoin d'une diversité de solutions.

une anticipation et une fluidité des règles législatives et réglementaires relatives à la mise sur le marché de ces produits. Ces derniers s'insèrent dans une réglementation européenne qui ignore la définition des produits de biocontrôle. Ce vide juridique rend le dispositif complexe et pose des difficultés d'interprétation entre les États membres. L'application de la réglementation est en conséquence peu lisible et affecte les évaluations et les autorisations de mise sur le marché, ainsi que le système de contrôle.

des agents de biocontrôle a été introduite dans la réglementation française en 2014. Cette définition indique que les agents de biocontrôle utilisent des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et qu'ils comprennent en particulier des macroorganismes, des microorganismes, des phéromones et des produits phytopharmaceutiques d'origine naturelle, qu'elle soit végétale, animale ou minérale. Les règles d'autorisation et d'utilisation en France de chacune de ces de chacune de ces catégories d'agents de biocontrôle sont parfaitement définies. Afin d'encourager le recours aux solutions de biocontrôle, l'État a prévu divers allégements, en particulier une réduction des délais et de la taxe d'évaluation. De plus, les produits de biocontrôle restent autorisés lorsque les produits conventionnels sont interdits, que ce soit dans les espaces verts ouverts au public, depuis le 1 janvier 2017, ou pour les jardiniers amateurs, à partir du 1 janvier 2019. La réglementation française encourage donc le recours aux produits de biocontrôle, qui concilient

à faible risque, les substances conventionnelles, les substances à substituer dès que possible et les substances à interdire. Elle ne prend pas en compte l'origine naturelle des substances ; cette lacune a été mise en évidence par l'évaluation de la réglementation européenne en cours. Le Gouvernement considère que le biocontrôle constitue, dans un certain nombre de situations, une alternative aux traitements chimiques conventionnels. D'ailleurs, le secteur du biocontrôle connaît en 2017 une croissance de plus de 25 %. Le plan Écophyto II +, que mes collègues et moi-même avons présenté le 27 juillet dernier, prévoit de nouvelles dispositions pour soutenir le développement du biocontrôle. La France défendra au niveau européen la promotion du biocontrôle et l'introduction d'une définition sein la réglementation européenne, notamment dans le cadre de la future révision du règlement (CE) n° 1107/2009 sur les produits phytopharmaceutiques. Cette vision est déjà partagée par un des colégislateurs : dans une résolution du 15 février 2017, le Parlement européen a souligné la nécessité de réviser

Une grande majorité d'entre eux sont assimilés à des agriculteurs du fait de leur affiliation à la mutualité sociale agricole, la MSA. Les autres dépendent du régime social de l'Établissement national des invalides de la marine, de par leur statut de marin pêcheur. veulent aujourd'hui voir leur profession reconnue statutairement comme une activité agricole pour une meilleure lisibilité juridique, sociale et fiscale. Ils pourraient alors relever à part entière des dispositifs rattachés, notamment au titre du régime des calamités agricoles et du regroupement en coopérative agricole. J'avais déposé

La pêche professionnelle en eau douce ne peut-elle être aujourd'hui considérée comme une activité agricole ? Je souhaiterais connaître votre intention, monsieur le ministre, concernant les revendications légitimes de ces professionnels.

le responsable d'une entreprise de pêche professionnelle en eau douce est considéré comme un chef d'exploitation agricole, une telle entreprise pouvant être assimilée à une exploitation piscicole, donc agricole, notamment du fait de la détention très fréquente des captures vivantes dans des viviers avant leur valorisation. En outre, les pêcheurs professionnels en eau douce sont affiliés à la MSA. Ils sont également soumis à la TVA agricole. La qualification de la pêche professionnelle en eau douce en tant qu'activité agricole n'a cependant jamais été explicite. jamais été explicite. L'action du Gouvernement sur ce sujet est simple. Aux fins de clarification définitive, et en vue d'éviter toute ambiguïté à l'avenir, la modification des articles L. 311-1 et L. 722-1 du code rural et

l'initiative de M. Bruno Retailleau, nous avons été nombreux à nous associer à la proposition de loi n° 508 du 12 avril 2017 tendant à reconnaître la saliculture comme activité agricole. Si l'exploitation du sel marin issu des marais salants est considérée comme une activité agricole dans de nombreux domaines- foncier, exploitation agricole, production, statut professionnel -, force est de reconnaître que les effets de la reconnaissance de la saliculture comme activité agricole sont assez divers, cette reconnaissance étant partielle En effet, la définition de l'activité agricole qui figure à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime fait actuellement obstacle à cette reconnaissance, alors que ce même code s'applique à cette activité et à ses producteurs. Les saliculteurs ne maîtrisent donc pas pleinement leur statut professionnel, faute d'avoir une connaissance complète de leurs droits et obligations. Monsieur le ministre, en février dernier, dans votre correspondance sur le statut des saliculteurs, vous m'indiquiez être prêt à soutenir les propositions législatives visant à simplifier et à mettre en cohérence la réglementation nationale.

Depuis plus de dix ans, les sauniers sollicitent une protection de l'appellation. Si cette décision de l'INAO devait être entérinée, elle mettrait à mal la démarche de spécialité traditionnelle garantie en cours et pourrait encourager concurrence déloyale et autres contrefaçons. En conséquence, monsieur le ministre, quelles réponses pouvez-vous nous apporter pour conforter le renouveau de la saliculture artisanale,

311-1 du code rural et de la pêche maritime sécuriserait la situation de fait des coopératives et des sociétés de forme agricole exerçant une activité salicole. Cette reconnaissance comme activité agricole n'aurait pas de conséquence de conséquence pour l'accès aux aides européennes, puisque le sel ne figure pas à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Outre une sécurisation juridique et une simplification pour les administrés, cette reconnaissance permettrait

Les zones de production de poires sont fortement touchées et, dans une moindre mesure, celles de pommes. Chaque année, de nouveaux foyers sont signalés en France comme chez nos voisins ; aucune région n'est épargnée. Actuellement, tout le matériel végétal est contaminé et peu de porte-greffes sont tolérants à la bactérie. Une journée chez les arboriculteurs du val de Durance a d'ailleurs été organisée la semaine dernière dans mon département des Hautes-Alpes ; le département voisin des Alpes-de-Haute-Provence est lui aussi affecté. Les dégâts sont importants, notamment sur les arbres qui ont été récemment renouvelés ; les jeunes vergers, de moins de cinq ans, et les arbres surgreffés semblent en effet plus vulnérables. C'est pourquoi la lutte contre le feu bactérien doit être traitée à la hauteur du danger qu'il représente pour la production française.

Les derniers essais prouvent que le BION 50 WG- fongicide qui induit une réaction de défense naturelle - est actuellement le produit le plus efficace. Il est autorisé en Europe, mais ne l'est pas en France.

la sénatrice Morhet-Richaud, le feu bactérien touche de façon cyclique les arbres fruitiers et ornementaux à pépins : pommiers, poiriers, néfliers et cognassiers. C'est un danger sanitaire de deuxième catégorie, pour lequel, selon l'importance et la configuration du foyer découvert, des mesures d'assainissement sont obligatoires, par la taille ou la destruction des végétaux. Ces mesures visent les pépinières, leur environnement et certaines zones de protection. Elles peuvent être étendues aux vergers de production par décision préfectorale. Le traitement de cette bactériose végétale est assez délicat et les produits actuellement autorisés ont une efficacité limitée. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a été saisi au printemps dernier d'une demande de dérogation visant à autoriser l'emploi du produit BION 50 WG pour la lutte contre le feu bactérien du pommier et du poirier. Ce produit est un stimulateur de la défense des plantes, autorisé sur cultures ornementales, sur le bananier et sur la tomate. Ce produit ne présente lui aussi qu'une efficacité partielle. Je vous rappelle que l'évaluation des substances se fait au niveau européen ; celle des produits

avant le 1 juin 2017 concernant le potentiel de perturbation endocrinienne de la substance. En parallèle, une demande d'autorisation pour l'utilisation du produit sur les pommiers et les poiriers a été déposée à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité

régulièrement pénalisés par les surtranspositions de textes européens. Monsieur le ministre, c'est un cri d'alarme que poussent les arboriculteurs de nos vergers alpins ! À ce jour, le travail de recherche, pourtant important, est insuffisant. Les investigations doivent s'intensifier afin de proposer aux arboriculteurs une sélection de matériel végétal très tolérant ou résistant à la bactérie, d'évaluer la sensibilité au feu bactérien du matériel végétal actuel, par variétés et porte-greffes,

Viticulture, polyculture, élevage sont terriblement affectés. J'appelle votre attention sur le fait que certains de ces territoires ont été frappés cinq fois de suite en cinq ans par différents sinistres. Par plusieurs courriers et contacts téléphoniques à votre ministère, j'ai déjà sollicité, en liaison avec les conseillers départementaux concernés, des mesures d'urgence.

De même, l'activation du fonds des calamités agricoles pour les pertes de fonds et les plantations se révèle indispensable. Par ailleurs, je signale que le chômage technique va frapper plusieurs exploitations. De surcroît, au regard

de 40 % à 60 %. Deuxième point, face à la multiplication des sinistres, en viticulture par exemple, il convient d'anticiper ces phénomènes par la mise en place de réserves dites « climatiques » consistant en un système de stockage du vin,

devrait, bien sûr, s'accompagner d'une fiscalité des stocks adaptée. Troisième point, compte tenu de la répétition des sinistres- cinq en cinq ans -, force est de constater, concernant les assurances, que la moyenne dite « olympique » ainsi que le seuil de déclenchement de l'indemnisation fixé à 30 % ne sont plus pertinents. Monsieur le ministre, comptez-vous mettre à l'étude, sans attendre, ces deux propositions majeures ?

des outils de gestion des risques adaptés. Vous l'avez rappelé, la filière viticole dispose d'outils spécifiques pour faire face aux aléas. Je pense au volume complémentaire individuel, qui permet de mobiliser les volumes mis en réserve les années précédentes pour combler le déficit de récolte de l'année, et aux achats de vendange, qui autorisent l'achat de raisins à d'autres producteurs pour compléter la récolte amoindrie sans changer de statut fiscal. Au-delà de ces dispositifs, les exploitants qui connaîtraient des difficultés peuvent également bénéficier du recours à l'activité partielle pour leurs salariés, d'un dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti pour les parcelles touchées par ces événements climatiques et d'un report du paiement des cotisations sociales auprès des caisses de la mutualité sociale agricole. Par ailleurs, il est indispensable que les agriculteurs puissent assurer plus largement leurs cultures à travers le dispositif d'assurance récolte contre les risques climatiques, incluant la grêle ou le gel, développé par l'État. Aujourd'hui, l'assurance récolte couvre 25 % des viticulteurs français. Pour soutenir son développement, les pouvoirs publics prennent en charge jusqu'à 65 % des primes d'assurance payées par les exploitants. Les producteurs ont aussi la possibilité de réduire le taux de franchise encore le seuil de déclenchement, afin de disposer d'un contrat d'assurance adapté à leurs besoins. Nous avons engagé des travaux avec la profession viticole et les assureurs pour faciliter une diffusion plus large de ce dispositif. Nous y travaillons avec les représentants des professionnels. Monsieur le sénateur, je vous rappelle que nous menons actuellement avec des députés et des sénateurs une réflexion sur des outils fiscaux permettant permettant notamment de travailler sur l'épargne de précaution ou la dotation pour aléas. Face à la multitude et à la multiplicité des risques climatiques auxquels nous devons faire face chaque année, je crois que ces mesures, qui seront discutées lors du prochain projet de loi de finances, seront les bienvenues.

l'alimentation. Monsieur le ministre, la carte des zones agricoles défavorisées, publiée le 28 mars dernier, a suscité de nombreuses réactions et questions, qui restent sans réponse à ce jour. elle conduit à l'exclusion de 230 exploitations sur quatorze communes situées dans le sud du département, pourtant inscrites dans le périmètre des zones humides d'importance au titre de la convention de Ramsar. Alors que le ministre de la transition écologique et solidaire envisage un nouveau plan Biodiversité, il paraît inconcevable et incompréhensible que ces espaces du marais poitevin ne soient plus considérés comme bénéficiaires de l'indemnité compensatoire des handicaps naturels. C'est un territoire exemplaire en matière de biodiversité et l'élevage est indispensable à l'équilibre écologique et économique de ces espaces remarquables. À ce titre, leur inscription est donc nécessaire, indispensable et souhaitée. le président du conseil départemental, Yves Auvinet, la présidente de l'association des maires et présidents de communautés de Vendée, Anne-Marie Coulon, les élus locaux, maires en tête, les agriculteurs et les parlementaires, dont Bruno Retailleau et moi-même très récemment, vous avons interpellé.

en Vendée. Le nouveau zonage, établi sur des critères nationaux, vise à garantir une homogénéité de traitement pour les agriculteurs, sous réserve de validation par la Commission européenne, ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui. Ces critères permettront de classer 14 210 communes, contre 10 429 dans le zonage actuel. Des paramètres complémentaires aux critères biophysiques ont été fixés pour confirmer que les territoires concernés n'avaient pas surmonté leurs handicaps et éviter ainsi les effets d'aubaine. Ce ciblage a été appliqué aux zones humides comme aux autres zones, ce qui explique la sortie du zonage des quelques communes du marais poitevin que vous mentionnez. Je mesure pleinement les difficultés et les enjeux que pose la sortie de l'ICHN pour les agriculteurs concernés. C'est pourquoi j'ai mis en place dès le 20 février dernier un dispositif d'accompagnement pour les agriculteurs sortant du zonage. Ce dispositif repose sur une sortie progressive des aides, comme le permet la réglementation européenne, la réalisation de diagnostics permettant d'identifier les opportunités de transformation pour ces zones autour de projets de filières. Je viens également d'ouvrir une aide permettant aux exploitations qui le souhaitent de réaliser un audit global et individualisé.

travailler avec l'ensemble des parlementaires, les présidents de conseils départementaux, c'est-à-dire l'ensemble des territoires, comme je l'ai déjà fait dans d'autres territoires où je me suis rendu, afin de trouver les solutions les plus adéquates

pêche maritime, modifié par la loi de 2005 relative au développement des territoires ruraux, précise que sont réputées agricoles « les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation Il s'agit des activités des entraîneurs de chevaux de course et des centres équestres qui étaient déjà, préalablement à cette loi, assujetties au versement des cotisations sociales des salariés auprès de la MSA. Elles sont classées dans la gestion de la MSA en référence au code accident du travail 150, sous l'appellation « haras, dressage, entraînement ». Ces différentes activités constituent trois branches professionnelles, dont les conventions collectives correspondent à des identifiants différents. la filière du cheval est confrontée à l'accélération de la procédure de restructuration des branches professionnelles mise en place par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et ce pour août 2018. La MSA a créé, au mois d'avril 2018, un service permettant aux employeurs de remplir leurs obligations vis-à-vis de la déclaration sociale nominative, avec production de bulletins de salaire. obligations et dispositifs futurs mettent en lumière des difficultés soulevées à plusieurs reprises par les organisations professionnelles auprès de vos services. D'une part, les secteurs sont répertoriés avec plusieurs dizaines de codes d'activité principale, d'autre part, les effectifs salariés sont comptés sous des appellations « haras » et « dressage » ne correspondant pas aux identifiants de convention collective. ministre, le règlement européen d'Eurostat définissant la méthode d'élaboration des statistiques agricoles européennes pour 2020 et les années suivantes ne mentionne pas, dans son projet d'évolution, les équins dans la liste des animaux devant être comptabilisés, alors qu'ils figuraient dans le précédent règlement. Monsieur le ministre, comment pensez-vous apporter aux entreprises de la filière les bases indispensables de classement de leurs différentes activités et de leurs emplois, mais aussi des statistiques européennes nécessaires pour élaborer une politique européenne du cheval dans le champ des activités agricoles ?

sur le premier point que vous avez soulevé, les différentes activités équines font l'objet d'une nomenclature variée, qui nuit à la lisibilité de l'ensemble. Sur la question des statistiques, la France avait demandé que les équins soient intégrés au projet de règlement, au même titre que les autres espèces animales de rente, ce qui,, n'a pas été retenu. viens à l'action du Gouvernement sur ce sujet. S'agissant des difficultés que rencontrent les acteurs de la filière équine dans le classement des activités et des emplois de ce secteur, un projet de nouvelle classification de ces activités au sein de la nomenclature des activités françaises a été proposé à la suite d'un travail entre le ministère de l'agriculture l'alimentation, les opérateurs et la MSA. Il va être soumis à l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui gère cette nomenclature. Par ailleurs, les partenaires sociaux des branches professionnelles des centres équestres et des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot et au galop sont pleinement engagés dans un processus de rapprochement de ces trois branches professionnelles. Comme vous le savez, ce rapprochement pourrait se traduire prochainement par la signature d'un accord collectif, ce que nous souhaitons. Au terme d'une période de cinq ans, une convention collective nationale couvrant ces différentes activités en remplacement des trois conventions qui existent actuellement pourrait être signée. Cette restructuration des branches professionnelles s'accompagnerait d'une réduction du nombre des identifiants des conventions collectives concernées. Enfin, sur la problématique des problématique des statistiques, en l'absence de reconnaissance à l'échelon européen, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation s'assurera que le cheptel et les activités équines restent bien à l'échelle nationale, notamment dans le cadre du recensement agricole, pour ce qui concerne les activités d'élevage. En effet, il importe que les équins, en tant que

Or ces métiers sont très peu valorisés et la profession fait face à un problème de recrutement. La pénibilité des tâches quotidiennes et les kilomètres parcourus représentent des difficultés pour les personnels. Il faut le reconnaître, ces métiers de service à la personne restent peu rémunérés et peu attrayants. Pourtant, ces emplois ne peuvent pas être délocalisés. Qui plus est, les besoins d'emploi deviennent de plus en plus importants avec le vieillissement de la population et la politique du maintien à domicile des personnes âgées. Pour rendre le métier un peu plus attractif, une revalorisation du point de salaire est nécessaire- l'indice n'a pas évolué depuis plusieurs années. La hausse du prix de l'essence rend également

nous faut également améliorer leur qualité de vie au travail. Pour faire face au vieillissement de la population et à l'augmentation des pathologies chroniques, il nous faut retravailler les référentiels d'activités, de compétences et de formation des aides-soignants ; ils seront revus d'ici au mois de mars 2019. L'objectif est de mieux tenir compte des spécificités de l'exercice des aides-soignants auprès des personnes âgées.

Prendre soin de ceux qui nous soignent », c'est également toute l'ambition de l'Observatoire national pour la qualité de vie au travail des professionnels de santé que j'ai installé au début du mois de juillet. Il concernera tous les professionnels de santé et médico-sociaux, qu'ils exercent en établissement, en ambulatoire ou à domicile.

100 millions d'euros seront consacrés à la réforme de la tarification de l'aide à domicile pour soutenir les acteurs et recruter du personnel. Monsieur le sénateur, au regard de ces différents éléments, je vous confirme qu'une offre de services de qualité reconnue, accessible et

Ces aidants à domicile sont formés ; 30 % d'entre eux ont un diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale. Pourtant, ils ne sont pas reconnus socialement ni financièrement. Leurs salaires sont extrêmement bas : les indices des grilles de début de carrière sont inférieurs au salaire minimum et les revalorisations acceptées par le ministère sont très faibles. Les indemnités de remboursement des déplacements restent bloquées à 0,35 euro par kilomètre depuis près de dix ans. Alors qu'une forte augmentation de l'activité de ce secteur est actuellement enregistrée, les structures, souvent associatives, ont de plus en plus de mal à recruter, en raison de la pénibilité du métier et des salaires indécents. Dans mon département, la fédération Aide à domicile en milieu rural, ADMR, de Haute-Loire représente

La situation est d'autant plus complexe que les conseils départementaux n'ont plus les capacités d'accroître leur soutien financier, dans la mesure où ils doivent déjà faire face à de nombreuses charges liées au vieillissement, à la dépendance, à l'aide sociale ou au handicap. Si aucune mesure n'est prise, des déserts des déserts de l'aide à domicile compléteront prochainement les déserts médicaux, alors que les besoins ne cessent d'augmenter. De plus, dans ce contexte, les personnes âgées et handicapées ne sont plus certaines de pouvoir accéder à des services de qualité à un coût supportable. Madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour répondre aux enjeux du vieillissement de la population et du financement de la perte d'autonomie ? Comment donnera-t-il les moyens nécessaires à ces salariés pour qu'ils remplissent pleinement leur rôle d'utilité sociale dans les meilleures conditions ? La parole est à Mme

dans les difficultés d'exercice. C'est pourquoi j'ai missionné la direction générale de la cohésion sociale pour définir et mettre en oeuvre des actions concrètes améliorant la qualité de vie au travail des professionnels du secteur médico-social. La commission Qualité de vie au travail dans les établissements et services médico-sociaux a proposé un plan d'action pour améliorer la qualité de vie au travail des professionnels en EHPAD. Les travaux de cette commission se poursuivront dès l'automne prochain pour les professionnels intervenant à domicile. En ce qui concerne les rémunérations- cela rejoint la question de M. le sénateur Jean-Claude Luche -, j'ai procédé à l'agrément par arrêté du 4 juin 2018 de l'avenant n° 36-2017 à la convention collective de la branche de l'aide à domicile, afin de mieux prendre en compte et rémunérer les temps et frais de déplacement des personnels effectuant des interventions occasionnant des interruptions d'horaires et des déplacements au cours de la journée. Cet accord aura un impact positif sur la rémunération des professionnels de cette branche. Des actions ont également été entreprises pour professionnaliser ces salariés et leur permettre d'avoir un parcours qualifiant, notamment avec la création du nouveau diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Par ailleurs, au-delà des différentes mesures évoquées, le Gouvernement entend mener une action en profondeur, afin de résoudre les difficultés structurelles des services d'aide et d'accompagnement à domicile et de permettre la modernisation de ce secteur. Nous le savons, les besoins vont considérablement augmenter. Un travail a été engagé pour rénover le mode de financement de ces services. Il sera accompagné d'une enveloppe de soutien de 100 millions d'euros en 2019 et 2020. Enfin, en lien en lien avec la feuille de route « grand âge et autonomie » que j'ai présentée lors d'une conférence de presse au mois de mai dernier, une réflexion plus globale sera conduite pour répondre au besoin accru de maintien à domicile et de coordination des acteurs

je vous remercie de cette réponse. L'aide à domicile peut permettre le développement de nombreux emplois, à condition, vous l'avez rappelé, que ces derniers soient attractifs. Nous devons impérativement et collectivement rechercher des solutions pour développer cette attractivité et permettre à nos aînés de bénéficier de la possibilité de rester à leur domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. La je souhaite vous alerter sur une situation inédite dans le sud du département de la Sarthe : depuis six mois, les femmes y sont dans l'impossibilité de réaliser une interruption volontaire de grossesse. En raison du départ à la retraite de l'un des médecins gynécologues, le centre hospitalier du Bailleul se trouve dans l'incapacité d'assurer ce droit essentiel pour les femmes, les praticiens restants faisant valoir leur clause de conscience spécifique concernant l'IVG, définie à l'article L. 2212-8 du code de la santé publique. Cet article dispose en effet que le « médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse ». Au mois de janvier 2017, le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes notait bien que, tant que cette clause de conscience demeurera, l'avortement ne sera pas un droit réel à part entière. Le cas sarthois démontre que, malgré les avancées obtenues durant le précédent quinquennat, notamment dans la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, dans la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ou encore dans la loi du 20 mars 2017 relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, le droit à l'avortement doit être conforté et assuré sur l'ensemble du territoire, afin que ce droit inaliénable soit pleinement reconnu. En ce mois de juillet, alors que Simone Veil est entrée au Panthéon, près de quarante-cinq ans après la reconnaissance du droit à l'avortement, il est intolérable que les femmes ne puissent pas exercer leurs droits essentiels, parce que des médecins, au mépris de l'accès aux soins, font valoir des réticences d'ordre personnel ou éthique.

Au regard de la situation sarthoise, quelles mesures envisagez-vous pour venir en aide aux femmes qui, depuis six mois, n'ont plus accès à un droit fondamental plus que jamais menacé et garantir ainsi l'effectivité de ce dernier ? La parole est à Mme la ministre

par ailleurs à vous assurer que mes services et l'agence régionale de santé, l'ARS, des Pays de la Loire se sont mobilisés, dès qu'ils ont eu connaissance de cette situation, en soutien de la direction de l'hôpital de Bailleul et des acteurs locaux, qui s'investissent aujourd'hui pour essayer de trouver une solution. La suspension de la pratique de l'interruption volontaire de grossesse au centre hospitalier de Bailleul est le résultat, vous le savez, de plusieurs facteurs : le départ à la retraite du praticien qui réalisait jusqu'à présent les IVG ; le recours à la clause de conscience des médecins encore présents ; une démographie médicale particulièrement affaiblie ces dernières années dans le département de la Sarthe. Face à cette impasse, la direction s'est assurée que les personnes concernées puissent trouver une réponse au centre hospitalier du Mans, situé à vingt-cinq minutes, et à celui d'Angers, également situé à vingt-cinq minutes, ces centres ayant des plages d'accueil et de soins réservées aux femmes qui en ont besoin.

accepterait de venir, à hauteur de 20 % de son temps de travail, au sein de cet hôpital. Si cette piste était confirmée, l'activité pourrait redémarrer au début du mois Par ailleurs, l'ARS a contacté l'hôpital du Mans, établissement support du groupement hospitalier de territoire, qui est prêt à soutenir, dans le cadre des axes du projet médical partagé, le centre hospitalier de Bailleul, au titre de la filière d'obstétrique.

défini entre les acteurs du territoire. Tout cela est en cours de négociation au sein de l'ARS. Le ministère suit avec la plus grande attention cette situation, accompagne et soutient les établissements de santé du département, dans cette dynamique territoriale, afin de répondre à ce besoin. La parole

En 2017, plus de 1 000 cas d'agressions ont été rapportés. Ce chiffre inquiétant ne peut qu'alerter, d'autant plus que certains professionnels ne déclarent pas les événements agressifs dont ils sont victimes, souvent par manque de temps, parfois par peur. de patients- pour une prise en charge qui ne leur convient pas, des prescriptions non conformes à leurs attentes, des temps d'attente jugés trop longs -entraîne insultes, menaces, harcèlement, vols, coups. Ces agressions se généralisent et suscitent un fort sentiment d'insécurité chez les praticiens. Les professionnels de santé, en premier lieu les femmes et les médecins généralistes, subissent une pression grandissante et avouent, pour certains, se sentir totalement démunis.

La médecine de proximité ne peut pâtir de telles difficultés et il ne faut en aucun cas aggraver les inégalités d'accès aux soins, d'ores et déjà criantes sur le territoire national. Madame la ministre,

Cette protection est primordiale pour leur assurer des conditions de travail décentes, sans lesquelles ils ne peuvent offrir des soins d'une qualité optimale à nos concitoyens. Les questions d'incivilité, voire de violence, que vous évoquez ne sont pas tolérables et je puis vous assurer que des mesures sont prises depuis plusieurs années par le ministère de la santé, en relation étroite avec les ministères de la justice et de l'intérieur. d'abord, l'ensemble des professionnels de santé bénéficient de dispositions pénales spécifiques leur offrant un régime de protection identique à celui de certaines fonctions et professions, comme les personnes investies d'un mandat électif public, les magistrats ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Les ordres professionnels de santé bénéficient également en vertu de la loi de certaines prérogatives de soutien à leurs membres. Les conseils nationaux, régionaux et départementaux des ordres peuvent par exemple exercer tous les droits réservés à la partie civile en cas de préjudice direct ou indirect à l'intérêt de leur profession, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'un de ces métiers. Au-delà de la protection pénale que je viens d'évoquer et du soutien, au besoin par la constitution de partie civile de l'ordre professionnel, il existe des séries de protocoles nationaux associant les ministères de la santé, de l'intérieur et de la justice, qu'il faudra certainement continuer à approfondir. Par ailleurs, cinq fiches réflexes du ministère de l'intérieur, mises à jour en 2017, délivrent une série de conseils pratiques sur la protection des professionnels de santé travaillant en secteur libéral et sur les réactions à avoir en cas d'agression. Enfin, depuis 2005, un membre du corps de conception et de direction de la police nationale est détaché auprès de la direction générale de l'offre de soins et a notamment en charge les questions d'incivilités et de violences.

Aujourd'hui, il importe de mieux former les médecins à la gestion des agressions verbales et physiques. Des méthodes se développent à l'hôpital, mais encore trop peu dans le cadre de l'exercice libéral. Il est vrai également que le déploiement du regroupement des professionnels de santé devrait atténuer la sensation d'insécurité. La parole

entre 1948 et 1977, et dont la toxicité est aujourd'hui avérée, a eu des conséquences délétères sur la santé de trois générations : elles-mêmes, leurs enfants et leurs petits-enfants.

le dispositif mis en place dans le cadre du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, comprenant la prise en charge intégrale de l'analyse du frottis par l'assurance maladie tous les trois ans, constituait une réponse adaptée aux risques auxquels sont exposées les « filles DES », victimes à leur tour du Distilbène. Or cette réponse ne convient pas, car elle méconnaît la nécessité du suivi spécifique de ces victimes, dont le risque de développer un cancer ACC du col utérin et du vagin est démultiplié.

constitue la condition indispensable d'une prévention pertinente pour elles. J'observe d'ailleurs que l'Institut national du cancer a précisé que les femmes sous traitement immunosuppresseur de longue durée, les femmes porteuses du virus de l'immunodéficience humaine et les femmes exposées au Distilbène présentaient un risque majoré de cancer du col de l'utérus et exigeaient un suivi spécialisé. Or, contrairement aux deux autres catégories de femmes que je viens de citer, les victimes du Distilbène ne bénéficient d'aucun statut particulier. De ce fait, elles ne sont pas incitées à effectuer un dépistage suffisamment régulier, eu égard à leur vulnérabilité spécifique. Cela peut constituer un risque majeur pour leur santé. C'est pourquoi je vous demande, madame la secrétaire

par le régime général d'assurance maladie d'une consultation gynécologique annuelle adaptée à leur situation et comprenant la réalisation d'un frottis spécifique ? La parole est à Mme la secrétaire

au nom de Mme Buzyn. Comme vous le savez, le Distilbène est un oestrogène de synthèse qui a été prescrit à partir des années 1940, vous l'avez rappelé, pour réduire le risque de fausse couche, et qui a été interdit en 1980, à la suite de diverses alertes sanitaires sur la nocivité du produit. Les femmes qui y ont été exposées sont confrontées à des anomalies du col de l'utérus et des trompes pouvant entraîner une stérilité ou des accidents de grossesse. Ainsi, depuis 2006, les femmes souffrant d'une grossesse pathologique liée à l'exposition au DES peuvent bénéficier d'un congé de maternité spécifique. Elles peuvent se voir attribuer le versement d'indemnités journalières maternité dès le premier jour de l'arrêt de travail et jusqu'au début du congé prénatal légal. Une telle prise en charge permet aujourd'hui de compenser la nécessité pour ces femmes de cesser le travail bien avant le début du congé prénatal. Ces femmes présentent également, et vous l'avez indiqué, un risque accru de développer certains cancers féminins. Le risque majoré de cancer du col de l'utérus a conduit l'Institut national du cancer à recommander un suivi particulier, avec la réalisation d'un frottis annuel. Le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus prévoit la prise en charge à 100 % d'un frottis pour les femmes n'en ayant pas réalisé lors des trois dernières années. L'arrêté qui définit le périmètre du dépistage précise bien que la deuxième génération des femmes exposées au Distilbène est incluse dans la population cible. Il est donc essentiel d'intégrer celles qui ne réalisent pas de frottis ou pas suffisamment régulièrement. assurées qui réalisent un frottis annuel, le frottis et la consultation, sans dépassements d'honoraires, sont intégralement pris en charge par l'assurance obligatoire et complémentaire dans le cadre des contrats responsables, lesquels représentent 95 % des contrats du marché.

que, entre le moment où la loi contenant cet amendement a été adoptée et le moment où les deux décrets d'application ont été publiés, il s'est passé quatre ans, six mois et quelques jours, ce qui est un sujet de réflexion

Je vous remercie

personnes handicapées. Madame la secrétaire d'État, le Président de la République s'était engagé, lors du débat du second tour de l'élection présidentielle, à créer « tous les postes d'auxiliaire de vie scolaire pour que les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l'école ». Il avait également promis de créer « les postes et les structures pour que les enfants, en particulier les jeunes autistes, n'aient plus à aller à l'étranger lorsqu'ils ont besoin d'aller en centre spécialisé En avril dernier, le Gouvernement a annoncé les mesures du quatrième plan Autisme mis en place sur cinq ans, notamment le triplement du nombre d'unités d'enseignement en maternelle, ces petites classes destinées aux enfants ayant besoin d'un soutien renforcé. De nouvelles classes spécialisées devaient également être ouvertes en primaire, au collège et au lycée. Une centaine de postes d'enseignants spécialisés dans l'autisme devaient être créés pour soutenir les enfants autistes accueillis dans ces classes. Au-delà de ces annonces, la réalité du quotidien des familles s'apparente chaque jour, et vous le savez, madame la secrétaire d'État, à un parcours du combattant. En effet, les budgets alloués aux ARS, qui font face à une recrudescence de la prévalence de ce handicap, limitent grandement les prises en charge. Les unités localisées pour l'inclusion scolaire diminuent chaque année le nombre de places disponibles pour les enfants atteints d'autisme ou ne renouvellent pas leurs autorisations de

Ces AVS sont pourtant essentiels pour les enfants en situation de handicap, singulièrement pour les enfants autistes. Ils leur permettent en effet de faire de grands progrès intellectuels et relationnels et connaissent, par leur formation, leurs besoins spécifiques. Madame la secrétaire d'État, les budgets alloués aux ARS, ainsi que le nombre de places adaptées à ces enfants, sont insuffisants et mettent les parents dans des situations de grande détresse. Au-delà, cette situation constitue une discrimination inacceptable en rompant avec le principe d'égalité scolaire. De nombreuses études démontrent que les troubles du spectre autistique constituent la maladie dont la prévalence a le plus progressé en trente En France, une personne sur cent est atteinte de trouble du spectre autistique, soit deux fois plus qu'aux États-Unis, et 60 % des enfants autistes ne sont pas scolarisés.

handicapées. Madame la sénatrice Perol-Dumont, la politique d'inclusion des personnes handicapées portée par le Gouvernement dans son ensemble entend ne laisser personne de côté. Les solutions doivent être bien sûr individualisées, adaptées à chacun, en fonction de ses besoins spécifiques. C'est dans ce cadre qu'agissent aujourd'hui les différents acteurs de l'accompagnement, avec le dispositif « Réponse accompagnée pour tous », qui se déploie massivement sur le territoire.

adoptée par le Gouvernement en avril dernier, bénéficie de 344 millions d'euros de mesures nouvelles, auxquels s'ajoutent 53 millions d'euros en provenance du troisième plan Autisme. Ces crédits serviront notamment

Je connais les difficultés des familles. Il s'agit de ne plus les ignorer et de veiller étroitement, avec les services, à trouver des réponses adaptées à ces situations individuelles. Ainsi, l'instruction diffusée aux ARS en mai 2017 impulsant l'évolution de l'offre sociale et médico-sociale pour personnes handicapées préserve le développement quantitatif de l'offre : 50 % des crédits y sont affectés, en priorité dans les zones en tension, là où il y avait un important retard de développement, pour faire face à des situations sans réponse et pour les handicaps les plus mal couverts et mal accompagnés. Pour la préparation des seconds projets régionaux de santé, j'ai également demandé aux ARS de veiller au développement de réponses mieux adaptées, notamment en réduisant de 20 % par an le nombre de personnes adultes

Madame la secrétaire d'État, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur la situation extrêmement préoccupante provoquée par la présence, à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France, de mineurs isolés étrangers, parfois très jeunes, en errance et refusant, malgré la forte implication de tous les acteurs depuis plusieurs mois, les prises en charge qui leur sont proposées. Parfois à la rue depuis leur plus jeune âge dans leur pays d'origine, le Maroc essentiellement, ces enfants commettent de nombreux actes de violence. Ils sont souvent devenus polytoxicomanes et se mêlent progressivement aux réseaux de délinquance organisée. Cette problématique concerne tout particulièrement le quartier de la Goutte d'Or, dans le XVIII arrondissement de Paris. Ces enfants et adolescents représentent un danger pour la sécurité des habitants et sont eux-mêmes en grand danger. La situation devient aujourd'hui d'autant plus alarmante que nous constatons tous l'impuissance des pouvoirs publics à répondre à la détresse de ces jeunes, qui sont à la fois victimes et délinquants. Or cette situation dépasse largement les compétences des collectivités locales en matière de protection de l'enfance. La coopération avec les autorités marocaines, mise en place depuis quelques semaines, mais qui ne semble pas être inscrite dans la durée, est un outil indispensable, ne serait-ce que pour permettre l'identification des jeunes. Néanmoins, elle ne saurait constituer la seule réponse à une situation qui relève d'abord de l'enfance en danger et de la protection de l'enfance et qui demande un engagement beaucoup plus fort des institutions qui en ont la responsabilité. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a écrit en ce sens au Premier ministre le 17 juillet dernier. Elle propose de travailler avec l'État à la création d'une structure adaptée à ces mineurs, qui fonctionnerait comme un centre éducatif fermé, en accordant une place prédominante aux soins. J'aimerais donc savoir, madame la secrétaire d'État, premièrement, quels moyens adaptés vont être déployés par l'État dans les mois qui viennent pour continuer d'activer les contacts diplomatiques avec les pays d'origine de ces mineurs isolés, en particulier le Maroc ; deuxièmement, pour renforcer les capacités d'action des forces de police dans les quartiers concernés ; troisièmement, pour trouver des réponses concrètes sur le plan pénal afin de sortir ces enfants de la rue et de leurs addictions,

La problématique des mineurs non accompagnés marocains mobilise fortement la justice, notamment les juridictions de la région parisienne, au premier rang desquelles le parquet des mineurs de Paris et le tribunal pour enfants. Vous l'avez dit, ces jeunes, souvent polytoxicomanes, vivent dans des conditions d'errance extrêmement précaires. Ils peuvent être à l'origine d'atteintes répétées à l'ordre public tout en étant eux-mêmes victimes de violences ou de réseaux de trafics. À Paris, il y aurait en permanence entre quarante et soixante-dix mineurs localisés dans le quartier de la Goutte d'Or, avec des arrivées et des départs continus. Ces mineurs représentent une part importante de l'activité de la permanence des mineurs du parquet de Paris. dernier, 813 mineurs ont été placés en garde à vue, dont 482 ont été déférés au parquet. Ces mineurs refusent en général les prises en charge et fuguent des dispositifs de placement. Les autorités françaises et marocaines unissent actuellement leurs efforts pour traiter la situation de ces mineurs non accompagnés, présumés marocains. Depuis le 18 juin dernier, les autorités marocaines ont dédié une mission, installée dans le commissariat du XVIII arrondissement, en charge d'identifier ces mineurs et d'établir leurs liens familiaux. Au cas par cas, des solutions seront apportées, dans leur intérêt et le respect de leurs droits. Dans ce cadre, les juges des enfants décideront de toute mesure adaptée. L'objectif est de sortir ces mineurs des rues et de les protéger. Nous souhaitons les inscrire dans un projet de réinsertion durable, familial et/ou institutionnel, tenant compte de leurs besoins fondamentaux en termes de santé physique et psychique et de leurs perspectives d'avenir, dans le cadre de la scolarité ou d'un apprentissage. Tous les acteurs compétents, français et marocains, travaillent en collaboration, dans le strict respect de la législation applicable. La parole

Les pouvoirs publics ne peuvent pas rester impuissants face à cette situation, qui nécessite de faire évoluer un certain nombre de méthodes et d'outils de travail concernant la justice des mineurs.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ma question porte sur le projet de construction d'un établissement pénitentiaire dans le Val-de-Marne. Mme la garde des sceaux avait annoncé, au mois de mars dernier, qu'une quinzaine de quartiers de préparation à la sortie seraient prochainement ouverts, sur le modèle des « prisons ouvertes » scandinaves. Je ne conteste pas l'objectif, à savoir mieux lutter contre la récidive, alors que plus 60 % des sortants de prison sont réincarcérés dans les cinq ans. Ce qui pose Ce qui pose question, c'est le choix de la localisation, tout particulièrement dans le Val-de-Marne, où deux emplacements sont envisagés. À Limeil-Brévannes, la construction d'une prison serait un coup dur porté aux projets de la ville, et ce pour deux raisons principales il y a déjà un projet de développement d'une zone d'attractivité économique sur la parcelle envisagée et la prison menacerait la construction de la future station de téléphérique des Temps durables. À Choisy-le-Roi, le site La construction d'un établissement pénitentiaire risque de freiner l'essor de la ZAC du quartier du Port. La ville de Choisy a besoin du développement de ces anciennes friches en bord de Seine, alors qu'elle souffre d'un réel déficit d'investissement en termes d'équipements publics. Surtout, je m'interroge sur le choix de construire un nouvel établissement dans le Val-de-Marne. La création de quartiers prioritaires de sécurité ne passe pas forcément par la construction de nouveaux sites. Elle peut passer aussi par des

la garde des sceaux a annoncé il y a un mois que le principe de la rénovation était retenu. C'est évidemment une bonne nouvelle. L'intégration d'un quartier de préparation à la sortie dans un centre pénitentiaire de Fresnes pleinement rénové apparaît aujourd'hui comme une éventualité. Ma question est donc simple et double : quels sont les projets de l'État pour la construction

Pour la seule Île-de-France, au regard des besoins projetés de la population pénale, ce sont six structures de ce type qu'il faut bâtir. Il s'agit d'établissements fermés, accueillant un public de personnes condamnées à de courtes peines ou d'autres, en fin de peine, dont le potentiel de réinsertion est avéré. la garde des sceaux vous sait gré de reconnaître l'opportunité de développer notre parc pénitentiaire en adaptant les structures aux différents types de publics qu'il doit accueillir. Elle regrette que vous considériez que ce nécessaire effort doit prendre place ailleurs que dans votre circonscription. Elle rappelle qu'une des réponses à la surpopulation carcérale forte que nous connaissons, au-delà de la refonte du dispositif de sanction et de l'échelle des peines qu'elle présentera dans le cadre du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, réside dans un programme immobilier ambitieux 15 000 places supplémentaires d'ici à 2027, dont 7 000 livrées à l'horizon de la fin de 2022. Limeil-Brévannes, au regard des propositions foncières qui nous ont été faites, est l'une des deux implantations envisagées pour le Val-de-Marne. Les études préliminaires montrent la faisabilité du projet, sans remettre en cause les perspectives de développement de la zone, particulièrement du projet de téléphérique urbain défendu par Mme le maire. Le choix d'implantation, comme pour l'ensemble du programme immobilier pénitentiaire et afin d'en garantir la cohérence, sera arrêté prochainement et en une seule fois. Les annonces correspondantes seront faites au moment de la présentation du projet de loi de programmation, au mois d'octobre. S'agissant, enfin, de la maison d'arrêt de Fresnes, Mme la garde des sceaux précise que des crédits d'étude ont été débloqués dès cette année afin de déterminer le programme de rénovation envisageable. La parole

La suppression annoncée du concours d'entrée en institut de formation en soins infirmiers au profit d'une sélection par Parcoursup dès le printemps 2019 suscite des inquiétudes. Ce processus de sélection, qui devrait ensuite être généralisé pour toutes les études paramédicales, nuirait notamment à la profession d'orthophoniste. Ces concours d'entrée en école d'orthophonie, difficiles mais essentiels, garantissent en effet une maîtrise de connaissances variées et nécessaires à cette profession. Ainsi, cette suppression risquerait d'entraîner un nivellement vers le bas, alors que la place des orthophonistes est amenée à croître, au regard notamment du vieillissement de la population. Enfin, il existe également un aspect économique, avec la mise en danger des établissements privés qui préparent à ces concours. Les supprimer brutalement, comme cela vient d'être fait pour les concours d'infirmiers, serait évidemment difficile pour leurs salariés.

Votre question porte sur les effets combinés de la mise en oeuvre de Parcoursup et du processus d'universitarisation des formations paramédicales sur l'accès aux formations en orthophonie. Agnès Buzyn et Frédérique Vidal ont conduit plusieurs cycles de discussion afin de dessiner les contours de la transformation des études de santé. C'est une nécessité afin de doter notre pays de professionnels de santé encore mieux formés et capables de s'adapter aux besoins croissants. L'universitarisation des formations paramédicales a vocation à rapprocher ces formations de l'université, afin de garantir les mêmes droits à tous les étudiants, tout en facilitant la transversalité et les approches interprofessionnelles entre futurs professionnels de la santé. Vous l'avez rappelé, les personnels soignants formés dans les instituts de formation en soins infirmiers seront admis sur dossier Parcoursup, et le profil de chaque candidat sera ainsi examiné pour ce qu'il est et non plus pour sa conformité avec les règles d'un concours. S'agissant des formations en orthophonie, la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants prévoit, conformément à un amendement adopté par le Sénat, que l'offre de formation disponible soit inscrite sur Parcoursup en perspective de la campagne d'affectation de 2019. Certaines formations pourront n'intégrer la plateforme qu'en 2020. L'intégration dans Parcoursup en tant que telle n'enlève rien au caractère sélectif de ces formations. La suppression de la hiérarchisation des voeux sur Parcoursup interdit les stratégies d'optimisation qui conduiraient certains à s'orienter en orthophonie « par défaut ». La spécificité de l'orthophonie sera ainsi respectée, ce qui n'enlève rien à la nécessité de réfléchir à la façon d'identifier plus finement les bacheliers ou les étudiants en réorientation qui correspondent le mieux aux attendus d'une formation en orthophonie. C'est ce à quoi le Gouvernement travaille en ce moment, en lien avec les écoles en orthophonie, les centres de préparation au concours et les professionnels du secteur. À ce stade, cette réflexion est toujours en cours, s'agissant tant du calendrier que des modalités d'accès aux écoles en orthophonie. Des annonces spécifiques auront lieu,

la secrétaire d'État, appeler votre attention sur les graves conséquences financières, pour les collectivités territoriales, qu'entraîne le retard chronique et systématique, en matière de notification, particulièrement, et de versement, par l'État, des subventions et des compensations financières et fiscales auxquelles elles ont droit. En dépit des nombreux engagements de l'État à ce sujet, ce problème récurrent n'a pas trouvé, à ce jour, de solution satisfaisante. Quelles que soient les règles en vigueur en matière de subventions et de compensations accordées par l'État aux collectivités locales, il doit pourtant être possible de définir et de mettre en oeuvre, de manière programmée et rigoureuse, une procédure qui permette, à terme, la notification et le versement intégral des dotations et des compensations avant une date limite précise. Pour mémoire, la liste des informations financières qui doivent être communiquées aux collectivités territoriales figure à l'article D. 1612-1 du code L'idéal en la matière serait que cette date tende à se rapprocher le plus possible du 31 mars, date limite prévue par la loi pour la communication des informations indispensables au vote du budget des collectivités. On ne peut sans cesse appeler à une gestion plus performante des collectivités locales si l'État ne fait pas preuve, de son côté, d'une véritable rigueur en matière de délais de notification, d'application et de versement des dotations et des compensations attribuées aux collectivités locales. À titre d'exemple, on peut citer le cas de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, notifiée en général aux mois de mai ou de juin, et pour laquelle les services de l'État exigent un commencement des travaux avant octobre de la même année Je vous demande donc quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour mettre en oeuvre, en étroite concertation avec les élus locaux, une procédure claire et rigoureuse et, surtout, un calendrier réaliste, particulièrement attendus par nos collègues élus en cette période d'austérité budgétaire. La parole auprès du ministre de l'économie et des finances. Madame la sénatrice Nadia Sollogoub, je vous réponds au nom du ministre de l'action et des comptes publics, dont je vous prie d'excuser l'absence. Vous interrogez le Gouvernement sur les délais de notification des dotations et des subventions allouées aux collectivités territoriales. Le respect de ce calendrier est une priorité pour le ministre de l'action et des comptes publics, tout comme d'ailleurs pour le ministre de l'intérieur, dont les services calculent et mettent en oeuvre les transferts financiers au profit des collectivités. Concernant les dotations et les compensations d'exonération, il s'agit d'informations indispensables pour que les collectivités puissent adopter leur budget dans les délais fixés par la loi, c'est-à-dire le 15 avril de l'année, au plus tard. Si la collectivité ne dispose pas, à la date du 31 mars, d'un certain nombre d'informations indispensables, le délai limite d'adoption de son budget est alors reporté. Par exemple, le calcul de la dotation globale de fonctionnement s'achève aux alentours du 31 mars, une fois que l'ensemble des données disponibles a pu être recensé et fiabilisé. Si la mise en ligne n'intervient pas le 31 mars, mais le 2 avril, alors le délai limite d'adoption du budget est reporté du 15 au 17 avril. La fin du mois de mars ou le début du mois d'avril sont des échéances incompressibles. Le recensement des attributions de compensation auprès des collectivités s'achève le 28 mars. Plus généralement, certaines données doivent, en vertu de la loi, provenir du dernier compte administratif disponible. Pour raccourcir les délais, il faudrait donc renoncer à utiliser les données de l'année écoulée et se fonder sur des données de l'année, C'est une éventualité que le Gouvernement exclut. En revanche, le ministère de l'action et des comptes publics ne partage pas votre observation relative aux subventions d'investissement, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de constater un « droit » pour la collectivité, mais bien de lui allouer une subvention sur la base des projets qu'elle aura proposés. Vous remarquerez d'ailleurs que la loi demande déjà au préfet de programmer la DETR avant le 31 mars. Soyez assurée, madame la sénatrice, que les services préfectoraux sont pleinement mobilisés, comme chaque année, pour examiner la trentaine de milliers de dossiers de subvention qui leur sont adressés aux mois de janvier et de février pour être en mesure d'effectuer une programmation rapide, judicieuse et efficace des crédits. La parole

supprimé 1 000 emplois et externalisé 85 % de ses activités clientèle, dont 30 % à l'étranger. Cette hémorragie s'est encore accélérée depuis deux ans par des délocalisations au Cameroun et au Sénégal, après le Maroc, le Portugal et l'île Maurice. Près de 3 000 emplois sont actuellement menacés par cette stratégie de délocalisation vers des pays à bas coûts de main-d'oeuvre. Ces délocalisations permettront des économies dérisoires, de l'ordre de 7 millions d'euros, à comparer au 1,4 milliard d'euros de bénéfices réalisés par le groupe en 2017, ceci dans le cadre d'un marché de 11 millions de clients générant 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. De surcroît, cette stratégie fait fi de la dimension humaine du sujet. Elle prévoit par exemple la formation du personnel à l'étranger par ceux-là mêmes qui, demain, verront leur emploi en France supprimé Ces milliers d'emplois sont pourtant souvent indispensables à l'économie locale française et à la cohésion des territoires. Certains de ces territoires seront considérablement affaiblis par la disparition des centres de « relation clients » et de leurs emplois. Lors d'une récente audition par la commission des affaires économiques du Sénat, Mme Isabelle Kocher, directrice générale d'Engie, a indiqué aux commissaires qu'« il n'y a pas d'avenir pour la relation clients ». déclaration, madame la secrétaire d'État ? Quelle appréciation l'État, actionnaire principal à hauteur de 24,1 % du capital et qui détient 28,1 % des droits de vote, porte-t-il sur cette stratégie d'entreprise ? Faut-il comprendre qu'Engie s'apprête à vendre ce portefeuille de 11 millions de clients dans le cadre, par exemple, de l'entrée de nouveaux partenaires au capital en compensation du retrait de l'État, comme pourrait le permettre le projet de loi relatif Enfin, quelles mesures l'État compte-t-il prendre pour préserver l'emploi de ces activités de relation clients en France et pour les relocaliser en France ? Bravo ! La parole est à Mme la secrétaire

dont l'État est l'actionnaire de référence. Sachez que nous sommes particulièrement attentifs à la dimension sociale de la transformation en cours de ce groupe. À cet égard, il faut signaler que le groupe a signé en avril 2016, avec trois fédérations syndicales européennes, un accord impliquant qu'une offre d'emploi au sein du groupe soit proposée à tout salarié concerné par des réorganisations. Cet accord prévoit, en outre, un important effort de formation. Sur le sujet spécifique du service client, la décision d'Engie d'externaliser une partie de son service résulte d'une intensification de la concurrence sur ses marchés, en lien avec la dérégulation des marchés de l'énergie. Le groupe a traversé une crise profonde jusqu'en 2016, à l'image des énergéticiens européens. Ces entreprises possédant un large portefeuille de clients sont confrontées à la nécessité de réduire leurs coûts, tout en proposant un service davantage en ligne avec les standards actuels, reposant sur les technologies numériques et une approche multicanale. Elles procèdent à une externalisation croissante des formes traditionnelles d'interaction avec la clientèle, éventuellement au travers d'opérateurs basés à l'étranger proposant des prestations moins onéreuses sur une plage calendaire et horaire élargie, et parallèlement au au déploiement d'outils avancés de CRM, ou, intégrant l'apport de nouvelles technologies faisant appel notamment à l'intelligence artificielle. Ce double mouvement d'externalisation des activités à faible valeur ajoutée et de recours croissant à des éditeurs de solutions et des entreprises de services numériques spécialisées s'inscrit dans la transformation numérique des processus. Les entreprises françaises spécialisées dans la relation clients tiennent donc, avec cette transformation, l'occasion de rebondir. Le groupe Engie a ainsi tout récemment confié à des sociétés françaises l'intégration de la relation clients numérique multicanale dans son système d'information. Dans ce contexte, les professionnels concernés et le Gouvernement travaillent au renforcement des atouts de nos entreprises et plus généralement à l'attractivité de notre pays. La parole

je constate que la question de la rentabilité du capital prime toute autre considération, et c'est bien dommage ! En réalité, l'État est aujourd'hui en situation de faire cesser les délocalisations

grandes entreprises ont signé avec le gouvernement italien un protocole limitant à 20 % les délocalisations des centres d'appels. Engie pourrait mettre en oeuvre en France un code de bonne conduite comparable, avec l'ensemble des acteurs

occupe ce que nous appelons la « Cité sanitaire » en partenariat avec la clinique mutualiste de l'Estuaire depuis 2012. Ce bâtiment est mis à sa disposition sous la forme d'un bail emphytéotique hospitalier. Ce montage juridique est, à ma connaissance, unique en France et n'a donc pas fait l'objet d'une réglementation spécifique. Aujourd'hui, le groupement de coopération sanitaire public de la Cité sanitaire se trouve dans une situation irrationnelle à l'égard de l'administration fiscale. En effet, celle-ci considère que ce groupement ne peut bénéficier d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en considérant qu'il n'est pas un établissement public de santé. Il en découle une taxation importante, d'un montant de 502 227 euros pour 2016 et de 533 149 euros pour 2017, à laquelle il convient d'ajouter 20 % de TVA. Pourtant, bien que le cas spécifique de la Cité sanitaire ne soit pas prévu par la loi, je considère que le groupement répond aux critères d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. l'immeuble est bien affecté à un service public d'intérêt général et le code général des impôts prévoit l'exonération des contrats de partenariat si le bien appartient à un établissement public ou est mis à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique hospitalier conclu avec un établissement public. En conséquence, je pense que ces éléments devraient être interprétés dans un sens favorable à la Cité sanitaire. Il faut également prendre en compte le fait que, si cet assujettissement devait prospérer, nous aboutirions au paiement d'une taxe foncière par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, qui serait sans doute l'un des seuls centres hospitaliers dans dans cette situation dans notre pays. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que le conseil municipal de Saint-Nazaire a voté, le 29 juin dernier, l'exonération de la taxe foncière du groupement de coopération sanitaire, comme le prévoit l'instruction fiscale de 2012. Le conseil départemental de Loire-Atlantique s'est engagé, pour ce qui le concerne, à voter une délibération identique, le 3 octobre prochain. Je souhaiterais donc, madame la secrétaire d'État, que vous me confirmiez la validité des décisions prises par les collectivités territoriales de la Loire-Atlantique, permettant ainsi la viabilité financière de la Cité sanitaire, dont les activités sont vitales pour nos concitoyens. La parole est à Mme la secrétaire auprès du ministre de l'économie et des finances. Monsieur le sénateur Yannick Vaugrenard, vous avez appelé mon attention sur la situation au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles construits dans le cadre d'un bail réel emphytéotique hospitalier conclu par le groupement de coopération sanitaire « Cité sanitaire nazairienne ». Les immeubles construits dans le cadre de tels contrats de bail sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant toute la durée du contrat. Cette exonération est soumise à plusieurs conditions. D'une part, pendant la durée du contrat, ils doivent être affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus pour la personne publique contractante. D'autre part, le bail doit avoir été conclu avec une personne publique visée au 1° de l'article 1382 du code général des impôts, ce qui inclut les établissements publics d'assistance dont font partie, selon la doctrine administrative, les établissements publics de santé. Enfin, à l'expiration du contrat, les immeubles doivent être incorporés au domaine de la personne publique contractante, conformément aux clauses de ce contrat. En application des dispositions de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, les groupements de coopération sanitaire sont qualifiés d'établissements publics de santé avec les droits et obligations y afférents. Lorsqu'ils sont érigés en établissements publics de santé par décision du directeur général de l'agence régionale de santé, ces groupements peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière. En revanche, les groupements qui n'ont pas le statut d'établissements publics de santé ne peuvent par définition pas bénéficier de cette exonération. En l'espèce, au vu des éléments à la disposition de l'administration fiscale, le groupement « Cité sanitaire de Saint-Nazaire » est un groupement de moyens constitué dans le but de réaliser et gérer la « Cité sanitaire ». Il ne bénéficie pas d'une autorisation d'activités de soins permettant de le qualifier, en application de l'article 6133-7 du code de la santé publique, d'établissement de santé. En conséquence, les bâtiments de la Cité sanitaire nazairienne ne peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière.

d'un partenariat public-privé. Nous connaissons les rapports de la Cour des comptes sur les partenariats publics-privés, notamment dans le domaine de la santé, qui sont interdits

Afin de le mettre en conformité avec la Charte de l'environnement, un chantier de réforme est aujourd'hui en cours. Le département de la Moselle, où de nombreuses mines ont été exploitées jusqu'au siècle passé, est directement concerné par cette réforme. Plus précisément, c'est le volet « arrêt définitif des travaux et après-mine » qui retient toute l'attention des Mosellans. À l'heure actuelle, comme vous le savez, madame la secrétaire d'État, c'est la loi du 30 mars 1999, dite loi après-mine, réformant le code minier, qui confie à l'État la prise en charge des problèmes posés par la cessation de l'exploitation minière, et ce au titre de la solidarité nationale. C'est ainsi que, pour l'essentiel, l'État est tenu de reprendre à sa charge les travaux d'entretien d'ouvrages de sécurité sur d'anciens sites miniers. Or, avec le dépôt à l'Assemblée nationale, le 23 novembre 2016, d'une proposition de loi, le projet de réforme du code minier est, de nouveau, d'actualité.

Elle prévoit, surtout, la création d'une mission d'indemnisation de l'après-mine. Examinée en séance publique les 24 et 25 janvier 2017 à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi est dorénavant en attente d'examen au Sénat. Pour autant, et parce que ce texte est de la plus haute importance pour tous les territoires qui ont connu l'exploitation minière, pourriez-vous d'ores et déjà me confirmer, madame la secrétaire d'État, que la mission d'indemnisation, dont la création est en soi une bonne chose, disposera bien de fonds

année, près de 40 millions d'euros sont ainsi consacrés par le ministère de la transition écologique et solidaire à la prévention des risques et à la réparation des dégâts miniers, au travers, notamment, de la surveillance des anciens sites miniers, de la réalisation de travaux de mise en sécurité et de l'indemnisation des dégâts miniers. Le code minier prévoit que l'exploitant minier reste responsable des dommages causés par son activité, et ce même après la fin de la validité de son titre minier. Il est donc tenu de réparer les dommages ou de les indemniser.

Depuis 2003, l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le FGAO, permet une préindemnisation, sous trois mois environ, à hauteur de 400 000 euros maximum, des particuliers dont la résidence principale est touchée par un dommage minier

Toutes les demandes d'indemnisation sont donc instruites avec un examen attentif permettant d'apporter des réponses au cas par cas. S'il n'existe pas, aujourd'hui, de mission d'indemnisation de l'après-mine, le de l'après-mine, le ministère indemnise déjà, directement ou par l'intermédiaire du FGAO, les victimes de dommages miniers et assume ainsi pleinement les obligations de l'État telles qu'elles lui sont fixées par la loi. Comme Comme indiqué dans la feuille de route de l'économie circulaire, portée par le ministère de la transition écologique et solidaire, le Gouvernement devrait engager la réforme du code minier à partir de la fin de cette année ou du Cette réforme est nécessaire pour permettre la valorisation des ressources minières françaises selon les meilleurs standards environnementaux et sociaux, comme vous-même l'avez souligné, monsieur le sénateur.

toute sa part au titre de la solidarité nationale en direction des populations concernées, qui vivent véritablement dans une angoisse de tous les instants. Sur le territoire

Cette angoisse appelle une réponse de l'État. J'ai bien noté les engagements que vous prenez et je me ferai fort de les répercuter sur le territoire en question.

l'Humanité aura consommé l'ensemble des ressources que la planète peut renouveler en une seule année. La quantité de carbone émise dépassera ce que nos océans et nos forêts peuvent absorber. M. le président Chirac disait, en 2002,

comme un désastre environnemental, écologique, social et économique, tel qu'on n'en a jamais connu en France

du Gouvernement. La France va d'ailleurs accueillir la prochaine réunion de l'IPBES, ainsi que, à Marseille, le congrès international de l'IUCN.

seules des exploitations exemplaires en termes environnementaux et socio-économiques [puissent] être envisagées en France ». Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, était en Guyane la semaine dernière pour faire un point de situation, alors que le débat public sur la construction de la mine vient juste de se terminer. Le rapport sera rendu public en septembre. Pour le Gouvernement, il était primordial que chacun puisse s'exprimer sur ce projet : les acteurs économiques, les ONG, les élus, mais aussi les représentants des peuples amérindiens. Le Gouvernement les a d'ailleurs rencontrés récemment. Je le sais ! En fonction des conclusions de ce rapport, la procédure prévoit que le porteur de projet apporte des améliorations significatives. Le Gouvernement n'a pas, pour l'instant,

je tiens à vous informer qu'une mission vient d'être lancée, avec le ministère de l'économie et des finances et le ministère des outre-mer, sur les enjeux socio-économiques et environnementaux des grands projets miniers en Guyane, en général.

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, quelques semaines après le vote de la loi relative à la SNCF, je crois indispensable d'alerter de nouveau le Gouvernement sur un aspect moins emblématique du réseau ferré national, celui des trains et, parmi ceux-ci, le POLT, le Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Le projet de TGV Limoges-Poitiers, promis à grand renfort de publicité et auquel ont été consacrés 150 millions d'euros dépensés en études, a fini par être enterré par le Conseil d'État, pour cause de non-financement. Pendant ce temps, la ligne POLT a été délaissée, avec le vieillissement de son matériel roulant, l'inconfort de ses voitures et ses retards fréquents, dus en partie à des locomotives tombant régulièrement en panne,

tout à la fois « structurante » et « prioritaire ». Je vous remercie donc, madame la secrétaire d'État, de faire savoir aux élus, aux chambres consulaires et aux forces vives des territoires concernés où en est la rénovation de cette ligne. Ma question se déclinera en cinq points.

le calendrier des travaux de régénération de l'ensemble de l'axe et de la mise en oeuvre du wifi, permettant aux usagers, notamment aux responsables d'entreprise, de communiquer ? Où en sont la commande des rames nouvelles 2022-2023 et la création d'un site de maintenance des enceintes ferroviaires à la gare de triage d'Estavel, à Brive ? Ces rames seront-elles bien adaptées à l'objectif de faire rouler ce train à 220 kilomètres à l'heure ? Est-il envisagé de rétablir le service quotidien d'un aller-retour sans arrêt entre Brive, Limoges et Paris ?

Dans la décennie à venir, cette ligne va bénéficier de très lourds investissements, pour régénérer l'infrastructure et renouveler le matériel roulant. En effet, d'ici à 2025, près de 1,6 milliard d'euros seront investis par SNCF Réseau dans la régénération de cet axe, afin de garantir la fiabilité du service rendu. Les investissements portent sur les voies et appareils de voies, la caténaire, la signalisation et les ouvrages d'art. Très concrètement, la régénération de la voie permettra de supprimer certaines limitations de vitesse et, ainsi, d'améliorer le temps de parcours. À ces travaux s'ajouteront un peu plus de 160 millions d'euros d'investissements déjà inscrits dans les contrats de plan 2015-2020 qui permettront d'améliorer la sécurité, la fiabilité et la régularité des trajets, grâce à la suppression de passages à niveau ou à la création d'installations permanentes de contresens. D'autres investissements complémentaires ont d'ores et déjà été identifiés, notamment la poursuite des relèvements de vitesse et le renforcement des installations fixes de traction électrique, en vue de renforcer la performance de la ligne.

Je concède que cette décision part d'une bonne intention, visant à mettre davantage l'accent sur l'évolution tendancielle et à lutter contre la volatilité des chiffres du chômage. Toutefois, le caractère tendanciel de ces chiffres peut être observé en continuant d'adopter une publication mensuelle et en étudiant les résultats avec une plus grande précision. Par ailleurs, ce temps de latence de trois mois empêche de calculer le taux de la population d'actifs dans le pays. Cela est dommageable, car, vous l'ignorez peut-être, bon nombre de nos voisins d'outre-Rhin continuent de publier les chiffres du chômage mensuellement, en rendant public le taux de la population active, afin d'escompter une action plus précise et coordonnée.

diffusent tous les trimestres, plutôt que mensuellement, comme auparavant, leur publication commune sur le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Ce rythme de diffusion est sans incidence sur celui de l'estimation des taux de chômage nationaux En effet, la publication trimestrielle Pôle emploi-DARES ne porte que sur les inscrits à Pôle emploi. Les chiffres concernant le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail et la population active continuent à être publiés par l'INSEE tous les trimestres. Par ailleurs, disposer d'une information mensuelle plutôt que trimestrielle sur les inscrits à Pôle emploi ne permet pas une analyse plus précise du marché du travail. En effet, les variations mensuelles du nombre de demandeurs d'emploi, à l'échelon national et, infranational, peuvent être fortement affectées par des phénomènes ne relevant pas directement de la conjoncture, tels que les comportements d'inscription sur les listes de Pôle emploi, la modification des règles d'inscription, ou encore l'indemnisation des demandeurs d'emploi. La parole

du ministère du travail. Néanmoins, il aurait tout de même été plus judicieux de prévoir une publication mensuelle, qui aurait permis d'adapter, au plus juste et en temps réel, l'ensemble des actions mises en oeuvre pour lutter contre le chômage. La parole

alors que le Gouvernement scande depuis plus d'un an que le travail et la lutte contre le chômage sont ses priorités- le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale du 4 juillet 2017, avait lancé : « Travaillons pour que le chômage reflue ! » -, les annonces concernant le futur budget pour 2019 sont sombres

sa suppression totale pour 2019 va entraîner des réductions de moyens et des fermetures de nombreuses maisons de l'emploi. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Sénat avait rejeté les crédits de la mission « Travail et emploi » lors de l'examen

La fracture numérique est de plus en plus flagrante et la dématérialisation des emplois et des offres est inaccessible pour ces populations. Les maisons de l'emploi ont un rôle important à jouer au quotidien, y compris pour favoriser l'accès à la mobilité l'aide à l'obtention du permis de conduire.

le chiffre de 4 000 suppressions d'emplois sur quatre ans étant évoqué par la presse. Or le chômage, après une légère baisse à la fin de l'année 2017, ne décroît pas de façon pérenne, à notre grand regret à tous.

Plusieurs opérateurs du service public de l'emploi sont notamment chargés de l'accompagnement des demandeurs d'emploi : Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi et l'APEC. La labellisation des maisons de l'emploi a en conséquence été arrêtée en 2009, et les missions ouvrant droit à un financement de l'État ont été progressivement concentrées sur deux axes l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ; deuxièmement, l'appui aux actions de développement local de l'emploi. En 2018, au vu des missions variables et très territorialisées des maisons de l'emploi et des besoins prioritaires incombant par ailleurs à la mission emploi », le choix a été fait, dans un contexte de contraction des finances publiques et dans la continuité des exercices budgétaires précédents, de poursuivre le retrait du financement de ces structures par l'État.

du PIC, ou plan d'investissement dans les compétences, notamment dans le cadre des appels à projets et expérimentations- formations aux métiers du numérique ou aux emplois verts, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, innovation, etc. Les pactes régionaux conclus entre l'État et les conseils régionaux seront également l'occasion de développer des actions de diagnostic des besoins en compétences des bassins d'emploi, domaine bien investi par les maisons de l'emploi. La parole est à M. Antoine Lefèvre,

Merci